Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, mesdames, messieurs, c’est avec stupéfaction et une tristesse immense que nous avons appris le décès de Didier Guillaume le 15 janvier dernier. Il est impossible d’évoquer la vie de Didier Guillaume sans rappeler son attachement à la Drôme et son parcours au sein du parti socialiste. Responsable départemental du mouvement des jeunes socialistes, Didier Guillaume s’engage au sein du comité de soutien drômois à François Mitterrand lors de l’élection présidentielle de 1981. Agent du Trésor public, il est élu pour la première fois conseiller municipal de Bourg de Péage en 1983. Il est directeur de cabinet du président du conseil général de la puis conseiller régional de Rhône Alpes en 1992. En 1995, il devient maire de Bourg de Péage, fonction qu’il occupera jusqu’en 2004,

se passionne pour l’agriculture et devient la même année conseiller politique de Jean Glavany, alors ministre de l’agriculture et de la pêche. Réélu conseiller général en 2004, il devient président du conseil général de la Drôme. Son arrivée au Sénat, en 2008, restera un moment privilégié de sa vie publique. Il défendra avec passion son département au sein de notre assemblée. Dès son arrivée au Palais du Luxembourg, il rejoint le groupe socialiste alors présidé par Jean Pierre Bel. Il sera successivement membre de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,

Au sein de la conférence des présidents, j’ai pu alors apprécier ses qualités humaines. En avril 2014, il succède à François Rebsamen à la présidence du groupe socialiste. La même année, il est rapporteur du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Son rapport concernant la modernisation des relations entre l’État et les fédérations sportives, remis en 2015, marquera notre assemblée. Membre de la délégation aux collectivités territoriales, il est rapporteur d’une mission d’information visant à rénover le dialogue entre l’État et les collectivités territoriales.

Le 16 octobre 2018, Didier Guillaume est nommé ministre de l’agriculture et de l’alimentation dans le gouvernement d’Édouard Philippe. Il s’implique notamment dans le dossier des pesticides et de l’épandage à proximité des lieux abritant des populations sensibles. Il est aussi attentif à la question du bien être animal. Le 10 juin 2024, Didier Guillaume est désigné par Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, Albert II, ministre d’État de la Principauté de Monaco, et met son engagement et ses compétences au service de la principauté. Passionné de politique, mais aussi de sport, et notamment de rugby, il aimait à citer Voltaire, pour qui « les passions sont les vents qui enflent les voiles du navire ; elles le submergent quelquefois, mais sans elles il ne pourrait voguer ». Didier Guillaume nous a quittés, et vogue désormais vers de nouveaux horizons. À ses anciens collègues, aux collègues de la Drôme d’aujourd’hui, Marie Pierre Monier, Gilbert Bouchet et Bernard Buis, j’exprime notre sympathie. À tous ceux qui l’ont connu au delà de cet hémicycle, j’adresse mes pensées.

Je vous remercie

Monsieur le Premier ministre, à la tristesse que vous avez exprimée et à la gratitude qui est la nôtre lorsque nous pensons à Didier Guillaume.

de la coupe du monde. Puis je rappeler qu’il était un amoureux de la côte basque et qu’il était passionné de Biarritz ? Cela nous a valu de partager de nombreux moments chaleureux.

une maladie foudroyante. Le Gouvernement est aux côtés du Sénat dans cette tristesse et dans cette gratitude.

la forte mobilisation, ainsi que celle des sénateurs membres de ce groupe, en faveur du renforcement des liens avec le Bundesrat. Cette visite revêt une portée particulière, puisque ce 22 janvier

J’ai moi même participé à Bonn, le 7 septembre dernier, au soixante quinzième anniversaire de la première session du Bundesrat, où j’ai eu l’honneur de prononcer une intervention solennelle sur la relation franco allemande.

Jean François Rapin, président de la commission des affaires européennes, ainsi que bien entendu Ronan Le Gleut et Audrey Linkenheld, respectivement président et secrétaire du groupe d’amitié Dans ces temps incertains pour la sécurité collective en Europe, dans l’attente des orientations qui présideront à la relation transatlantique et alors que plusieurs États membres de l’Union européenne traversent des turbulences politiques, le couple franco allemand conserve plus que jamais sa pertinence. La diplomatie parlementaire y a toute sa part. Mes chers collègues, en votre nom à tous, je souhaite à Mme la présidente Anke Rehlinger la plus cordiale bienvenue au Sénat de la République française ! L’ordre

Alors que je vous alertais sur les conséquences de votre politique libérale orthodoxe, dont l’alpha et l’oméga sont la réduction continue de la dépense publique, et donc la destruction du service public, vous m’avez répondu avec un aplomb certain

face à l’épidémie de grippe ? Sont elles imputables, selon vous, à l’inefficacité du personnel ? Monsieur le Premier ministre, vous qui fûtes ministre de l’éducation nationale, ne constatez vous pas les défaillances actuelles de notre système éducatif :

J’ai souri en vous entendant dire que nous menions une politique libérale effrénée… « Orthodoxe » ! Je vous propose de communiquer votre intervention à divers organes de presse qui ne semblent pas partager exactement votre vision… Je voudrais simplement vous rappeler les efforts que nous avons faits dans ce budget en faveur du service public. Dans le domaine de l’éducation, j’ai souhaité que nous abandonnions la proposition du gouvernement de mon prédécesseur Michel Barnier visant à supprimer

Ce climato sceptique, qui avait qualifié, à l’époque, le réchauffement climatique de « canular », tourne le dos, pour la seconde fois, au reste du monde, dans le combat contre le dérèglement climatique. Les dramatiques incendies de Los Angeles n’ont pas modifié son analyse.

décision et pour éviter que ce club des quatre ne grossisse ses rangs à l’avenir

la décision des États Unis de sortir de l’accord de Paris et de se retirer de l’Organisation mondiale de la santé. Je tiens à vous

Cet effet de « cocotte minute » se traduit par une augmentation significative de la violence : plus de 50 % des infractions pénales commises à Mayotte le sont par des personnes en situation irrégulière. La situation est dramatique. Encore aujourd’hui, des échauffourées ont eu lieu entre la population et les migrants.

On ne reconstruira pas Mayotte si l’on n’apporte pas des solutions concrètes et très fermes pour faire face à l’immigration illégale. Cela suppose une volonté,

Lors de votre premier déplacement dans vos nouvelles fonctions, au centre pénitentiaire de Liancourt, vous avez exprimé votre préoccupation face à ce qu’il faut bien appeler la crise de notre système carcéral. Le plan « 15 000 places », qui visait à créer 15 000 places de prison supplémentaires se voulait une réponse massive, pragmatique, à ce problème. Or notre taux d’incarcération continue d’augmenter.

de faire son autocritique et de revoir sa copie. Les attaques envers les bureaux et les agents de l’OFB sont inacceptables. Les critiques des plus hauts responsables politiques, en pleine élection des chambres d’agriculture, ne sont pas non plus de nature à apaiser les débats, alors que certains syndicats se chargent déjà d’attiser les braises d’une situation hautement inflammable. Doit on rappeler que la police de l’environnement est une chance vu les bouleversements climatiques que nous connaissons ? Le président Trump a déjà fait sortir son pays de l’accord de Paris, alors que les incendies les plus dévastateurs de l’histoire de la Californie ont ravagé 16 000 hectares depuis le 7 janvier Nous devons rester fermes sur la défense de l’environnement et soutenir les agents qui assurent ces missions essentielles. Madame la ministre, puisqu’il est de bon ton de critiquer de plus en plus ouvertement l’OFB, pouvez vous nous dire si ses missions sont remises en cause ? Le cas échéant, qui les assurera demain ?

en agriculture permettra de simplifier certains régimes de sanctions. Il s’agit d’aller directement à la sanction administrative, de façon à proportionner les contrôles

Il nous faut maintenant travailler à rassembler. Les équipes du Premier ministre recevront la direction de l’OFB et les organisations syndicales, ce vendredi. Vous pouvez compter sur nous pour continuer à soutenir haut et fort les missions de l’OFB, en pleine intelligence avec les personnes La parole est à M. Patrick Kanner, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

au Parlement un texte sur la taxation des hauts patrimoines ? Allez vous imposer aux salariés 7 heures de travail non rémunérées ? Renoncerez vous à diminuer l’indemnité journalière des fonctionnaires en cas d’arrêt maladie ?

Monsieur le président Kanner,

Monsieur le ministre, la lutte contre le narcotrafic et la criminalité est un combat national dont vous vous êtes emparé avec la volonté de réarmer l’État. La responsabilité de ce dernier est lourde, mais la part incombant aux communes n’en est pas moins importante. En effet, il est de la responsabilité des maires de protéger les habitants

sur l’État ? Pouvons nous collectivement mener ce combat essentiel à l’avenir de la France si certains refusent de s’y associer ? Bref, quelle réflexion pouvons nous engager sur ce sujet sans remettre en cause le principe de la libre administration des collectivités territoriales ?

Le 21 janvier dernier, les résultats balistiques ont permis de faire le rapprochement précis entre ces deux faits. D’autres tirs sont survenus la même nuit dans une autre commune, notamment contre contre un commerce. La gérante a indiqué que son mari, actuellement incarcéré pour association de malfaiteurs, devait passer en jugement le 21 janvier. Elle supposait elle même l’existence d’un lien avec les violences du 18 janvier dernier.

pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. L’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche est une source d’inquiétude pour nous, Européens, et fait peser de sérieuses menaces sur les relations transatlantiques et les équilibres commerciaux mondiaux.

carbonée. Dans ce nouveau contexte, comment le Gouvernement, aux côtés de ses partenaires européens, entend il se positionner pour être le moteur d’un commerce international équilibré et respectueux de l’accord de Paris ?

Grâce à l’impulsion donnée par le Président de la République depuis 2017, l’Europe dispose de tous les outils pour se défendre contre les pressions commerciales, soutenir notre industrie et assurer notre souveraineté numérique.

L’Union européenne doit aussi faire un effort spécifique pour améliorer sa compétitivité et développer de nouveaux partenariats. Nous ne sommes pas opposés par principe aux accords commerciaux ; nous regardons au cas par cas le résultat des négociations, en fonction de nos intérêts.

de l’accord de Paris et proposer l’augmentation des importations de gaz issu de fracturation hydraulique repousse les limites du « en même temps ». Alors que tous les capitaux américains, publics et privés, vont être au service de l’administration Trump Musk, les exportations et la compétitivité de la France de demain sont assurées par les investissements d’aujourd’hui. Cette semaine, votre gouvernement, soutenu par la majorité sénatoriale, a raboté les crédits consacrés au plan France 2030, aux universités

Monsieur le ministre de l’intérieur, ma collègue Marie Mercier et moi même souhaitons vous interroger sur les violences urbaines qui ont embrasé ce week end le quartier des Saugeraies à Mâcon, en Saône et Loire. Trois bâtiments communaux sportifs ou sociaux ont été détruits, en plus de véhicules incendiés, et les forces de police ont été attirées dans de véritables guets apens. Les dégâts sont estimés à plus de 1 million d’euros. d’euros. Ces émeutes exaspèrent la population ; ces attaques contre nos biens communs révoltent leurs usagers ; ces dégradations désespèrent le contribuable. D’autant plus que les précédentes émeutes de l’été 2023 ont laissé la ville de Mâcon sans solution satisfaisante pour assurer ses bâtiments communaux, les franchises dépassant désormais 2 millions d’euros par site. Aux dires du préfet de Saône et Loire et du maire de Mâcon, notre ancien collègue Jean Patrick Courtois, ces actes interviennent sur fond de narcotrafic. Les tags retrouvés à proximité des événements sont explicites « Donnez nous un local, ou c’est la guerre ! », pouvait on lire. Dans notre pays, les dealers en sont donc à exiger des locaux communaux pour se livrer à leur commerce et embraser un quartier face à la résistance courageuse et légitime des pouvoirs publics. Au delà des propositions sénatoriales pertinentes défendues par nos collègues Étienne Blanc et Jérôme Durain, comment comptez vous réarmer notre République pour ne pas perdre la bataille de la confiance de nos concitoyens, et surtout gagner la guerre contre le narcotrafic ?

monsieur le ministre. Je souhaite m’associer à l’hommage que vous avez rendu aux forces de sécurité ; la coopération a été parfaite entre les policiers, les gendarmes, les sapeurs pompiers, mais également entre les services de la préfecture et la procureure de la République.

Ces phénomènes climatiques représentent une menace croissante pour les infrastructures publiques. Or de plus en plus de collectivités se trouvent aujourd’hui dans l’incapacité de souscrire un contrat les primes d’assurance contre les risques climatiques, qui ont en moyenne augmenté de 90 % entre 2024 et 2025, ont atteint des niveaux prohibitifs pour plus de 1 500 communes. Les conséquences d’une telle augmentation sont désastreuses pour nos collectivités. Plusieurs d’entre elles se retrouvent exclues du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (CatNat), qui constitue pourtant l’ultime rempart contre les aléas climatiques. Nos territoires d’outre mer se trouvent en première ligne face aux effets du dérèglement climatique. L’intensité des cyclones atteint désormais des niveaux records. Le territoire métropolitain n’est pas en reste : le 1 janvier dernier, le maire de Breil sur Roya a dénoncé par l’absurde l’incapacité à assurer sa commune en interdisant par arrêté les catastrophes naturelles sur son territoire. Si cet exemple prête à sourire ou à pleurer, il traduit en creux l’effondrement du principe de socialisation des risques, pourtant au fondement de nos régimes d’indemnisation.

votre question porte sur les difficultés que rencontrent certaines collectivités territoriales pour s’assurer face aux risques climatiques. Ces difficultés sont réelles ; j’ai pu le constater sur le terrain à la suite des inondations qui se sont produites dans le Pas de Calais entre novembre 2023 et janvier 2024.

annulé unilatéralement par son assureur en 2024. Ces situations ne sont pas acceptables et interrogent sur le mode de fonctionnement du régime assurantiel applicable

l’adaptation au changement climatique, est également renforcé. J’invite les collectivités qui ne trouvent pas d’assureurs à se rapprocher du bureau central de tarification (BCT), soit l’autorité administrative chargée de garantir l’accès aux assurances obligatoires. C’est lui qui a permis de débloquer la situation à Breil sur Roya,

Ils sont exaspérés, car ils voient se répéter des comportements qui bafouent nos lois, menacent notre sécurité et piétinent notre souveraineté. Désormais, ils attendent des actes forts. Les appels à la haine, à la violence et au meurtre diffusés par certains influenceurs algériens résidant en France ne sont pas de simples provocations : ce sont des actes de déstabilisation, une menace directe pour notre sécurité intérieure. Ces individus qui prospèrent sur notre sol, tout en sapant nos valeurs, incarnent une cinquième colonne que nous ne devons plus tolérer.

plus fortement. Ma question est simple : quelles seront vos prochaines mesures pour éradiquer ces menaces ? Envisagez vous de prendre de nouvelles décisions : suspendre la délivrance de visas ou dénoncer, voire rompre, les accords de 1968 ?

Amazon a t il menti sur son offre initiale ? Le Gouvernement a t il menti devant la représentation nationale ? J’attends de vous que vous puissiez nous éclairer à de rappeler les épisodes précédents. Il y a dix mois, lors des questions d’actualité au Gouvernement, j’interrogeais votre prédécesseure sur la volonté d’EDF de confier à Amazon l’hébergement des données relatives au renouvellement des pièces de nos centrales nucléaires.

Or la presse nous apprenait récemment que ladite expérimentation avait pris fin, faute d’avoir obtenu d’Amazon la garantie que les données seraient hébergées en France et ne seraient pas transmissibles à des services américains. Lesdites données étaient donc bien sensibles.

La parole est à M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

et sécurisée. Pour les données non sensibles, de grands acteurs internationaux proposent des services à des prix compétitifs et à des conditions techniques extrêmement exigeantes, utilisés par un certain nombre d’acteurs publics et privés. Les données sur lesquelles EDF travaille avec Amazon dans le projet que vous citez portent sur des informations non sensibles, pour lesquelles le risque que vous évoquez n’existe pas.

le procureur de la République, les caisses d’allocations familiales, les caisses primaires d’assurance maladie, ainsi que les forces de gendarmerie et de police qui, grâce à de petites équipes de cyberenquêteurs,

deuxièmement, le soutien à une meilleure efficience du service public de l’eau ; troisièmement, la garantie d’une évolution contenue des prix pour le consommateur.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

et de la loi du 23 juillet 2010 prise pour son application, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis favorable sur la nomination de M. Laurent Hénart dans les fonctions de président du conseil d’administration de Voies navigables de France.

afin de pouvoir passer à l’examen de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». À défaut, nous devrons reporter l’examen des amendements restants à la fin des missions ce soir. Il nous reste vingt six amendements à examiner.

Cet amendement a pour objet, à périmètre constant, de geler, au niveau fixé en loi de finances initiale pour 2024, la dotation globale des autorités administratives indépendantes rattachées au programme 308 « Protection des droits et libertés » au titre de leur participation

de 3,1 % en euros constants avec correction de l’inflation. Cette diminution est toutefois inégalement répartie entre les deux programmes de la mission. Le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » concentre en effet l’essentiel de la baisse des dotations en crédits de paiement. À l’inverse, le programme 308 « Protection des droits et libertés » connaît une hausse en crédits de paiement

j’avais indiqué que l’effort pouvait difficilement porter sur les autorités administratives indépendantes. Au delà d’un certain nombre de projets spécifiques tels que le déménagement dans de nouveaux locaux

ancien Premier ministre coûte 200 000 euros de frais de déplacement et de secrétariat à la République. C’est absolument inacceptable pour la France qui travaille.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c’est seul que j’ai l’honneur d’ouvrir cette année l’examen en séance publique de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Éric Bocquet, avec qui j’avais commencé l’examen de ce budget et dont je tiens à saluer les travaux, a quitté le Sénat le 1 novembre 2024. Pierre Barros, qui l’a remplacé pour achever cet examen, est absent pour motif familial impérieux, et nous lui adressons une pensée amicale. Je serai donc bref. Les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » demandés pour 2025 s’élèvent à 30,4 milliards d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Au premier abord, il s’agit d’une légère diminution, de 2,3 %, par rapport à la loi de finances initiale pour 2024. Cette baisse résulte toutefois d’une mesure de périmètre, le programme support des ministères sociaux ayant été transféré de la mission « Solidarité, insertion et égalité Les crédits alloués à chacun des trois autres programmes augmentent en réalité de 2,12 % par rapport à 2024. Cette hausse des dépenses s’explique par le

En revanche, à rebours de la tendance récente à la mobilisation de la prime d’activité pour soutenir le pouvoir d’achat, les crédits qui sont dédiés à la prime d’activité diminueraient en 2025 de 1,5 %, à hauteur de 10,3 Le Gouvernement a déposé un amendement visant à diminuer les crédits de la prime d’activité de 91 millions d’euros supplémentaires. La commission a rendu un avis de sagesse, qui pourra être bienveillante, madame la ministre,

à la partie valeur, si je puis le dire ainsi ? Quelles modifications envisagez vous dans le calcul de la mesure ? Comment fixerez vous les paramètres ? Et quelle sera votre philosophie en la matière ? Nous avons besoin d’être éclairés sur ces points. Le contexte dans lequel s’inscrit ce budget a incité la commission à se montrer défavorable à la grande majorité des initiatives visant à augmenter les crédits de la mission, d’autant plus qu’il s’agit de l’une des missions les mieux préservées par les efforts de redressement des comptes publics. À titre d’exemple, les crédits pour l’aide alimentaire augmentent dans le projet de loi de finances pour 2025 de 3,4 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2024. Les nouveaux moyens alloués en 2025 permettront notamment la mise en œuvre d’actions portant sur l’alimentation des très jeunes enfants ou encore la montée en charge du programme Mieux manger pour tous (MMPT), qui cherche à faire rimer aide alimentaire et qualité nutritionnelle, et qui est très apprécié par les associations. De même, les crédits destinés à financer la politique d’égalité entre les femmes et les hommes augmentent de 10 % entre la loi de finances initiale Comme l’année précédente, l’augmentation des crédits constatée est entièrement absorbée par la mise en œuvre de l’aide exceptionnelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, versée en une fois dans un délai de trois à cinq jours aux femmes qui quittent leur foyer pour fuir leur conjoint violent. La budgétisation initiale de cette prestation pour 2024, fixée à 13 millions d’euros, s’est révélée largement insuffisante, comme nous le prévoyions l’an dernier, puisque l’exécution de 2024 s’est établie à 26 millions d’euros, soit le double. le projet de loi de finances prévoit 20 millions d’euros pour cette aide, dans l’hypothèse d’un taux de recours stabilisé. Compte tenu des contraintes budgétaires et de la relative préservation de la mission « Solidarité,

services d’aide par le travail (Ésat). En effet, ces structures médico sociales, qui sont déjà largement en déficit, ne pourront pas dans leur grande majorité absorber cette nouvelle dépense. Plusieurs amendements visent à faire financer par l’État une partie de la part de l’employeur. La commission y est favorable et appellera à les voter. Nous aurons également un débat sur la prise en charge de la prime Ségur dans les organismes de la branche sanitaire et sociale, ce qui nous donnera l’occasion de demander au Gouvernement de préciser ses intentions, son chiffrage du besoin et son appréciation de la situation financière des associations qui mettent en œuvre ces politiques. Je vous inviterai donc, mes chers collègues, à adopter les crédits de la mission ainsi modifiés.

les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » traduisent une ambition forte en faveur de l’inclusion sociale et de l’égalité, et sont le reflet d’un engagement politique au service des plus vulnérables. À ce titre, il faut souligner qu’il s’agit de l’une des rares missions qui, dans un contexte budgétaire plus contraint que jamais, connaît une augmentation de ses moyens de plus de 2 % par rapport à l’année 2024. Dans ce contexte, la commission des affaires sociales a soutenu, dans son ensemble, la répartition des crédits de la mission. Cependant, lors de son examen des nombreuses politiques publiques financées par cette mission, la commission a soulevé deux points d’attention sur lesquels je voudrais revenir.

concerne les crédits alloués au programme 157 « Handicap et dépendance », nous tenons à saluer les mesures prises depuis plusieurs années en faveur d’un rapprochement des droits des travailleurs protégés et des travailleurs en milieu ordinaire, notamment dans les Ésat. Cependant ce rapprochement ne peut se faire Cependant ce rapprochement ne peut se faire indéfiniment au prix de la stabilité financière de ces établissements. C’est pourquoi nous proposerons de compenser la moitié du coût de l’obligation de mise en place d’une complémentaire santé dans les Ésat, soit 18 millions d’euros, afin de les soutenir dans l’attente d’une réforme structurelle de leur modèle de financement. Cela nous semble d’autant plus nécessaire que l’État s’y était engagé. Enfin, sur un enjeu qui concerne l’ensemble des programmes de la mission, la commission s’inquiète des conséquences pour le secteur associatif et les collectivités territoriales de l’extension, en juin dernier, par la ministre du travail, de deux accords de la branche associative, sanitaire, sociale et médico sociale Ces accords permettent à l’ensemble des salariés de la branche de bénéficier des mesures du Ségur – soit 238 euros brut mensuels – et s’appliquent de manière rétroactive au 1 janvier 2024. Il faut se féliciter de cette avancée au profit du pouvoir d’achat des salariés. cette mesure n’a fait l’objet d’aucun abondement des dotations dont bénéficient associations et collectivités, conduisant à des situations financières dégradées pour ces dernières. Il nous semble qu’il y a, là encore, une réflexion à mener dans les mois à venir afin de pérenniser les acteurs de la solidarité dans nos territoires.

! Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps de l’intervention générale et celui de l’explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes pour intervenir.

la crise est l’occasion de se rappeler l’importance de la solidarité et de l’entraide » : ces mots de Nelson Mandela résonnent avec force en ce moment, dans un contexte instable, incertain et tempétueux. Cette crise nous confronte surtout à une réalité incontournable : la solidarité ne doit pas devenir une variable d’ajustement budgétaire et encore moins la victime de l’instabilité gouvernementale, mais doit plutôt en être le pilier. Le contexte particulier qui nous occupe, marqué par l’absence de budget adopté au 1 janvier, est particulièrement inquiétant. Cette mission, qui totalise près de 6 % des crédits de paiement du budget général, est cruciale pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables pour lesquelles les errances budgétaires peuvent avoir des effets majeurs. Ces populations méritent au moins la stabilité et au mieux un soutien accru. La loi spéciale permet déjà la stabilité, c’est un moindre mal. Pour 2025, l’effort en faveur de la mission semble maintenu, ce qui est à saluer. Toutefois, plusieurs points d’alerte persistent et je souhaite les aborder aujourd’hui après avoir remercié nos collègues rapporteurs Arnaud Bazin et Laurent Burgoa pour leurs travaux sur les crédits de la mission. Cette mission représente en 2025 un montant total de 30,37 milliards d’euros, soit une hausse des crédits à périmètre constant de 2,13 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2024. L’augmentation permet de compenser, dans une certaine mesure, l’inflation et les revalorisations successives des prestations, notamment pour la prime d’activité et l’allocation aux adultes handicapés, qui représentent désormais 81 % des crédits de la mission. Mais derrière cette stabilité, se cachent des difficultés, en particulier pour les départements, et c’est là un point majeur de notre préoccupation quant à cette mission. En effet, malgré les avertissements que nous avions lancés l’année dernière, force est de constater que la situation des départements reste particulièrement fragile. Nous avions notamment lancé l’alerte sur la compensation des frais relatifs à la mise à l’abri et à l’évaluation des mineurs non accompagnés (MNA), or nous craignons que la situation ne persiste en 2025.

Cette absence de compensation intégrale des dépenses est par ailleurs alourdie, cette année, par les coûts liés à l’extension des mesures du Ségur. En effet, les accords signés le 18 juin dernier pour étendre les mesures du Ségur à l’ensemble des salariés du secteur médico social prévoient une revalorisation salariale de 238 euros brut mensuels, rétroactive au 1 janvier 2024. Cette mesure représente un coût supplémentaire de 600 millions d’euros, répartis entre la sécurité sociale, l’État et les départements. Si cette avancée a été largement saluée par les acteurs du secteur, nous regrettons qu’aucun abondement des dotations n’ait été prévu pour compenser cette charge. Les départements se voient là encore contraints d’assumer cette revalorisation salariale sans soutien financier de l’État.

situation de handicap. Il a permis des progrès notables, notamment en posant les bases d’une accessibilité universelle, en instituant le droit à compensation pour les surcoûts liés au handicap et en renforçant l’inclusion scolaire. Ces avancées méritent d’être saluées, et nous nous félicitons notamment de de voir désormais quatre fois plus d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire par rapport à 2006. Cependant, le bilan reste encore largement perfectible et nos travaux sur le budget pour

Nous regrettons que de nombreuses avancées obtenues il y a vingt ans dans la loi ne se concrétisent pas aujourd’hui dans les faits. Ce constat, mes chers collègues, nous rappelle l’importance de notre mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques.

Ces structures jouent un rôle fondamental dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, mais leur situation devient de plus en plus incertaine. Les crédits alloués à ces établissements connaissent une légère baisse en 2025, alors que les coûts d’adaptation, notamment la mise en place d’une complémentaire santé pour les travailleurs handicapés, continuent d’augmenter à hauteur de 338 euros par travailleur. Cette situation met en péril la pérennité des Ésat et leur capacité à remplir leur mission d’insertion. La mission couvre également des enjeux essentiels tels que la petite enfance. La réforme du service public de la petite enfance (SPPE) est une ambition légitime pour améliorer l’accès à l’accueil des jeunes enfants. Toutefois, la mise en place de cette réforme soulève des interrogations concernant sa compensation financière, notamment pour les intercommunalités. Le financement de 86 millions d’euros prévu pour 2025 ne devrait pas suffire à compenser les coûts réels liés à cette réforme, et la lisibilité de son application reste incertaine pour de nombreuses collectivités. Madame la ministre, mes chers collègues, face à ces défis et malgré leurs alertes, les élus du groupe Union Centriste s’engagent à soutenir ce projet de loi de finances, en espérant vivement que les questions soulevées dans le cadre de nos débats seront prises en compte, en particulier pour ce qui est des départements et du soutien renforcé

Cette situation saugrenue, voire ubuesque, ferait presque oublier que, entre temps, le Président de la République Emmanuel Macron a perdu les élections européennes et les élections législatives, et que le gouvernement de Michel Barnier est tombé à défaut d’une majorité à l’Assemblée nationale.

Malheureusement, rien n’a changé en matière de politique sociale depuis un an. Quelque 2 000 enfants dorment toujours dans la rue. Les inégalités sociales entre les plus riches et les plus précaires n’ont jamais été aussi criantes. Les étudiantes et les étudiants font la queue devant les banques alimentaires. Et des millions de familles peuvent basculer dans la précarité ou la grande précarité du jour au lendemain. De plus, à l’heure de célébrer les 20 ans de la loi de 2005 sur le handicap, de nombreuses entreprises continuent de préférer payer une amende plutôt que d’embaucher des personnes en situation de handicap et l’obligation d’accessibilité des espaces publics n’est toujours pas entièrement respectée. Pis encore, le Gouvernement ponctionne 50 millions d’euros sur le budget de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph),

leur montant n’est toujours pas à la hauteur. Le Gouvernement se félicite de la hausse des crédits en faveur de lutte contre les violences faites aux femmes, mais les chiffres sont têtus. Le PLF pour 2025 prévoit 85 millions d’euros quand il en faudrait au moins 2,6 milliards et que le coût total des inégalités entre les femmes et les hommes est évalué à 118 milliards d’euros par an… Nous ne sommes clairement pas sur la bonne échelle d’investissement. Ce PLF prévoit également la montée en charge du dispositif de l’aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales. Je rappelle que ma collègue Michelle Gréaume a été à l’initiative de cette proposition.

L’État doit tendre la main à ces victimes et les aider à franchir le cap, mais le montant moyen des aides universelles d’urgence versé jusqu’à présent ne dépasse pas 864 euros,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous étudions une mission dont le périmètre est plus lisible que les années précédentes, car il a été recentré sur les seuls programmes d’intervention. programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » a été rattaché à une autre mission et nous gagnons en cohérence. Cette mission essentiellement sociale est confrontée, malheureusement, à des besoins en augmentation et les crédits alloués, en particulier ceux qui sont attribués au programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes », ne prennent pas la mesure des politiques publiques nécessaires pour répondre durablement aux problèmes posés. C’est notamment le cas pour le Pacte des solidarités, lancé à la fin de 2023 pour remplacer la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Le collectif Alerte qui rassemble trente sept fédérations, associations nationales et collectifs interassociatifs locaux de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, l’avait qualifié l’année dernière de « pauvre plan contre la pauvreté ». Il déplore cette année que « le compte n’y soit toujours pas ». Selon les derniers chiffres de l’Insee, le taux de pauvreté des enfants de moins de 18 ans est plus élevé de six points que celui de l’ensemble de la population. Un enfant sur cinq est désormais concerné et 8 millions d’enfants vivent dans des ménages dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Nous avons besoin de réformes structurelles pour endiguer la pauvreté, à tous les âges de la vie et ce, dès la naissance. Nous approuvons l’augmentation des crédits alloués au programme Mieux manger pour tous, mais la dynamique des besoins la rend toujours insuffisante. insuffisante. Les associations d’aide alimentaire restent préoccupées quant à leur capacité à remplir leurs missions dans un contexte de forte hausse et d’intensification de la précarité, alors que certains approvisionnements diminuent et que les prix alimentaires sont durablement élevés.

Victor Hugo, qui a siégé dans cet hémicycle, écrivait que « ceux qui ont faim ont droit ». Il est temps de constitutionnaliser le droit à l’alimentation et de le rendre effectif. C’est l’objet d’une proposition de loi que le groupe écologiste a déposée l’année dernière.

cette année encore, les augmentations de crédits prévues dans cette mission sont en trompe l’œil. En effet, le nombre des bénéficiaires des programmes de solidarité, d’insertion et d’égalité des chances augmente de sorte que les dépenses devraient suivre. le Gouvernement propose simplement le maintien des moyens qui, en plus d’être insuffisants, ont subi l’inflation. Plus de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Ce sont souvent des femmes seules avec leurs enfants, des travailleurs pauvres, des retraités et des personnes en situation de handicap.

Les Ésat participent au financement des moyens de transport, des complémentaires santé et de la restauration des travailleurs et travailleuses, mais ces dépenses nouvelles ne doivent pas conduire à fragiliser leur budget.

Enfin, dans le programme 157, il est important de rétablir le maintien de l’AAH pour les bénéficiaires qui exercent un travail à temps partiel, au delà de 50 %. qui est du programme 137, les crédits pour l’égalité entre les femmes et les hommes augmentent. Malheureusement, le nombre de femmes victimes de violences qui doivent être accompagnées augmente aussi dans des proportions bien plus élevées. Le Gouvernement a enfin accédé aux demandes visant à étendre les revalorisations Ségur aux centres d’information

d’une augmentation sensible, de 4,8 %, due essentiellement à sa déconjugalisation. Je souhaite d’emblée revenir sur la question de l’extension des mesures

Toutefois, certaines associations, notamment celles qui accompagnent les victimes de violences conjugales, n’ont pas perçu de crédits pour financer la prime

autre sujet : les difficultés des départements à prendre en charge les mineurs non accompagnés. Beaucoup d’entre eux sont totalement dépassés par la situation, et les 101 millions

La solidarité et l’égalité des chances sont des principes fondamentaux qui font la force de notre République et qui nous renvoient à l’une de nos valeurs essentielles : la fraternité. Il nous faut tout faire pour préserver notre système de solidarité sur le long terme, même si cela n’exclut pas de surveiller les dépenses et l’efficacité des mesures dans tous les domaines.

Si j’approuve totalement la ligne budgétaire stricte, fixée par le Gouvernement et soutenue par mon groupe, je suis également sensible à la protection des plus vulnérables et à la question cruciale de l’accès aux droits. Dans cet esprit, je souhaite évoquer l’expérimentation en cours du préremplissage des déclarations trimestrielles de ressources pour les allocataires du RSA et les bénéficiaires de la prime d’activité, dans laquelle se sont engagés cinq départements, dont le département des Alpes Maritimes. Cette expérimentation vise plusieurs objectifs : fluidifier et faciliter les démarches administratives, réduire les tâches chronophages et les erreurs, sécuriser les données.

cette expérimentation a plusieurs effets positifs. Tout d’abord, c’est une réussite sur le plan technique, puisque le préremplissage s’est déroulé sans embûches par une connexion et un partage de données entre plus de 10 000 employeurs, auxquels s’ajoutent les partenaires associés et organismes sociaux.

Enfin, il est prévu, à terme, que le préremplissage des déclarations contribue à un allégement des tâches chronophages avec, pour corollaire, un repositionnement des équipes sur l’accompagnement des usagers les plus fragiles, ce qui est véritablement nécessaire.

La seconde a trait au « porté à connaissance » de ce dispositif lorsqu’il sera généralisé à ceux qui, bien qu’ayant des droits à exercer, ne le sollicitent pas. Au niveau national, le taux de non recours est de 34 % pour le RSA

à l’heure où de nombreuses démarches sont dématérialisées et où, selon l’Insee, près de 17 % d’entre nous sont encore mal à l’aise avec les usages du numérique.

Cela montre combien toutes nos actions sont complémentaires. Enfin, je ferai une ultime observation. Il existe actuellement des bases de ressources différentes selon les prestations sociales versées, ce qui se traduit, pour une même famille, par des règles différentes de prise en compte des types de ressources, ou de périodicité des calculs, selon les prestations qu’elle perçoit. Il semble par conséquent indispensable, pour s’inscrire dans une vision globale, de long terme,

Ensemble, nous nous sommes donné pour cap de soutenir nos services publics, tout en réduisant la dépense publique. Tenir ce cap relève de notre devoir, celui de sauvegarder notre modèle social français, auquel nous avons toutes les raisons d’être tant attachés ! La parole

la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » représente à elle seule près de 6 % des crédits inscrits dans le présent projet de loi de finances. Elle participe activement, en complément du projet de loi de financement de la sécurité sociale, à la préservation de notre modèle social. En 2025, ses crédits s’établiront à plus de 30 milliards d’euros, en hausse de 2,13 % à périmètre constant – cet effort doit être souligné dans le contexte budgétaire contraint que nous connaissons. Ils permettront de poursuivre les politiques menées ces dernières années en matière de lutte contre la pauvreté, d’inclusion des personnes vulnérables et de renforcement de l’égalité des droits. Le programme 157 « Handicap et dépendance », dont les crédits s’établissent, pour 2025, à près de 16 milliards d’euros, en hausse de 4,22 %, promeut une société plus inclusive, garante de l’émancipation individuelle des personnes handicapées. La quasi totalité de ces crédits sont dédiés au financement de l’allocation aux adultes handicapés dont la forte augmentation s’explique par la hausse du nombre de bénéficiaires et les effets de la déconjugalisation pour quelque 120 000 bénéficiaires. Je me réjouis du succès de cette réforme que nous sommes nombreux à avoir soutenu sur ces travées. En 2025, des mesures bienvenues d’harmonisation du calcul de l’AAH bénéficieront aux salariés travaillant dans les établissements et services d’aide par le travail ou en milieu ordinaire. Ces avancées s’inscrivent dans un contexte de rapprochement des droits sociaux de leurs travailleurs du droit des salariés en milieu ordinaire, même si cela soulève des inquiétudes sur la pérennité du financement de ces structures. Le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » connaît une relative stabilité de ses crédits qui s’élèvent, en 2025, à 14,26 milliards d’euros. Ce programme retrace les très nombreuses politiques menées par le Gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté et de protection des personnes vulnérables. Il assure principalement le financement de la prime d’activité, du revenu de solidarité active, en outre mer et dans les départements où il a été recentralisé, et de la prime de fin d’année attribuée aux ménages les plus fragiles. La baisse limitée des crédits de ce programme s’explique à la fois par la stagnation du nombre de bénéficiaires de la prime d’activité et par la mise en œuvre progressive de la réforme de la solidarité à la source, conformément à l’engagement du Président de la République. Cette réforme, qui tend à lutter contre le non recours aux prestations sociales, mais également contre les risques d’indus, se poursuivra en 2025. En matière de protection de l’enfance, ce budget prévoit une hausse de la compensation aux départements de la mise à l’abri des mineurs non accompagnés et du financement des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Cette compensation demeure cependant limitée pour des départements qui font face à une hausse continue de leurs dépenses. Je salue aussi la mise en place, dans le cadre de la mise en œuvre du service public de la petite enfance, d’un accompagnement financier des communes et des intercommunalités qui se sont vu confier le rôle d’autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant. Le programme 304 comporte également les crédits destinés à lutter contre la précarité alimentaire. Ils connaîtront en 2024 une hausse de près de 2 %. Au niveau national, le ralentissement de l’inflation devrait donner un peu d’oxygène aux banques alimentaires, mais la vie chère en outre mer appelle plus que jamais la mise en œuvre de politiques spécifiques. et les hommes » retrace une partie des crédits destinés à améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes. La hausse de près de 10 % de ses crédits par rapport à 2024 s’explique principalement par le recours à l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales. Rappelons que les crédits alloués à cette politique interministérielle atteignent 5,78 milliards d’euros, une enveloppe en nette augmentation depuis cinq ans.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » reflète l’engagement de notre République envers les plus vulnérables.

Les crises successives ont exacerbé les inégalités et rendu plus visibles encore les défis auxquels nous devons faire face. Dans un contexte budgétaire pourtant contraint, ce projet de loi de finances se caractérise Tout d’abord, le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », avec une dotation de 14,26 milliards d’euros, demeure un levier essentiel pour soutenir les ménages modestes et encourager l’activité professionnelle. La prime d’activité, principal poste de ce programme, continue de jouer un rôle crucial, avec un budget d’un peu plus de 10 milliards d’euros. Toutefois, la légère baisse de ses crédits, bien que cohérente avec une diminution prévue du nombre de ses bénéficiaires, appelle une vigilance accrue face aux effets de l’inflation sur le pouvoir d’achat des travailleurs précaires, précaires, d’autant que le Gouvernement nous proposera tout à l’heure de diminuer les crédits de la mission de près de 92 millions d’euros… Nous notons également une augmentation des crédits pour l’aide alimentaire, qui témoignent de la nécessité d’un engagement continu envers les personnes les plus vulnérables, même s’il faut s’inquiéter du profil émergent des personnes qui en bénéficient : de plus en plus de jeunes enfants et d’étudiants. S’agissant du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes », nous nous réjouissons de la progression de 10 % des crédits, une hausse essentiellement due au financement accru de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales,

Depuis le début de l’année, six femmes – déjà ! – ont été victimes de féminicides en France. Six vies brisées, six drames qui rappellent tragiquement l’ampleur de ces violences. Derrière ces chiffres se cachent des histoires de souffrance, des appels à l’aide trop souvent restés sans réponse. Ces actes barbares constituent une atteinte intolérable à la dignité humaine et traduisent une faillite collective, alors même que nous avons Nous ne pouvons plus tolérer que des femmes meurent sous les coups de ceux qui prétendaient les aimer. Face à cette urgence, il est impératif de renforcer les dispositifs de prévention, d’écoute et de protection des victimes, et de mobiliser tous les moyens nécessaires pour que ces femmes puissent se libérer de l’emprise de leurs bourreaux. Enfin, le pacte des solidarités, outil stratégique pour lutter contre la pauvreté, voit son budget augmenter de 23,4 %. Les mesures phares telles que les petits déjeuners à l’école, la tarification sociale des cantines, ou encore le fonds d’innovation pour la petite enfance témoignent d’une volonté claire d’agir dès le plus jeune âge pour prévenir les inégalités. Cependant, des inquiétudes persistent. Nos collectivités locales, en première ligne de la mise en œuvre de ces politiques, connaissent des difficultés croissantes, notamment face à l’inflation qui pèse sur les coûts de la restauration scolaire. Avant de conclure, je souhaiterais saluer l’engagement des associations et des bénévoles qui se battent au quotidien contre ces inégalités et apportent leur soutien aux plus vulnérables.

J’ai eu l’honneur de recueillir le soutien du Sénat, l’an dernier, sur un amendement du groupe socialiste qui visait à augmenter de 2 millions d’euros le budget du Crédit national des épiceries sociales (Cnes). Nous nous félicitons que cette hausse ait été pérennisée.

Il s’agit d’un signal plus qu’alarmant. Concernant la protection des enfants et des jeunes vulnérables, je rappelle que le nombre d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance a augmenté de près d’un quart en six ans. Et pourtant, beaucoup ne sont pas encore protégés et les drames se succèdent.

Si les dépenses des départements pour assurer l’accueil, le séjour et l’hébergement des enfants à protéger ont explosé ces trois dernières années, la solidarité nationale, elle, n’est pas à la hauteur, puisque les crédits sont en recul et, au mieux, stagnent. Dans le même temps, le Gouvernement opère un prélèvement sur les finances départementales, amoindri, mais bien réel, au titre de l’ancien fonds de précaution. Concernant les jeunes majeurs de moins de 21 ans sortant de l’ASE, la compensation qui sera accordée par l’État aux départements s’élève à 50 millions d’euros, soit le même montant cette année qu’en 2024, alors que les exécutifs départementaux nous signalent l’augmentation de ces dépenses et que, en parallèle, les crédits dédiés à la stratégie nationale de protection de l’enfance sont en baisse de 14 %. Il n’y a donc aucune nouvelle réjouissante pour ces enfants et pour celles et ceux qui les accompagnent, ce qui n’est pas acceptable. Aussi, nous avons déposé un amendement visant à financer un plan d’urgence pour les pouponnières – l’urgence dans l’urgence ! La commission d’enquête de nos collègues députés est catégorique : la situation est plus qu’alarmante,

je veux rappeler que le pessimiste voit dans toute opportunité une difficulté supplémentaire, quand l’optimiste voit dans toute difficulté une opportunité. Je veux faire le choix de l’optimisme : faisons de cette difficulté budgétaire – car, disons le, le budget de cette mission n’est pas à la hauteur – une opportunité, celle de réaffirmer collectivement qu’il faut aller plus loin et ne pas fléchir !

Mais les chiffres ne doivent pas masquer une réalité vécue par de très nombreux concitoyens confrontés à des difficultés grandissantes. Mon propos portera sur le programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes », dont le budget est en hausse de 10 % par rapport à l’an passé. Cette augmentation couvre en grande partie l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, qui est en hausse de 7 millions d’euros. L’aide universelle d’urgence est une avancée législative importante, qui résulte, je le rappelle, d’une proposition de loi sénatoriale, dont je tiens à saluer l’auteure, notre ancienne collègue et désormais ministre, Valérie Létard. Encourager à porter plainte, mettre en place les conditions pour inciter les femmes à quitter le domicile, tel est l’objet même de cette aide financière. L’argent ne doit plus être un frein pour les victimes. Si nous saluons un budget en hausse, il est toutefois difficile de se réjouir d’une augmentation des crédits, laquelle traduit la hausse des besoins des victimes, toujours plus nombreuses, et reflète autant de situations de détresse pour elles et leurs enfants. En huit mois, plus de 26 000 personnes auraient bénéficié de l’aide universelle d’urgence. Je rejoins le rapporteur spécial : la réussite de ce nouveau dispositif tient en partie au rôle d’accompagnement du secteur associatif. Je salue et remercie l’ensemble des personnels qui œuvrent en leur sein. Nous connaissons les efforts qu’ils consentent pour écouter, orienter, accompagner et contribuer à ce que toute violence soit dénoncée. Nous sommes nombreux à saluer le travail des associations d’aides aux victimes, ainsi que des centres d’information sur les droits des femmes et des familles.

Nous mesurons la nécessité d’avoir des personnels formés et un accompagnement social et psychologique durable, mais aussi l’impérieuse nécessité d’une coordination entre les différents acteurs.

Mais, en 2025, la violence à l’égard des femmes est et reste un véritable fléau dans notre société. Le combattre nécessite la mobilisation de tout un chacun, citoyens, associations, acteurs judiciaires. Permettez moi d’espérer que, à l’avenir, nous aurons davantage de lisibilité, à la hauteur de ces enjeux, et non une succession de dispositifs éparpillés entre différentes missions budgétaires. Nous sommes le vingt deuxième jour de l’année et six femmes ont déjà été tuées par leur conjoint, tandis que des milliers d’entre elles continuent à appeler à l’aide, parfois, malheureusement, dans un parfait silence. Depuis 2017, cette lutte est une grande cause nationale. Certes, des évolutions législatives ont eu lieu et sont à souligner. D’un point de vue juridique, je pense au bracelet antirapprochement, au téléphone grave danger, récemment aux ordonnances de protection immédiate. D’un point de vue civil, j’ai à l’esprit la question du recouvrement des pensions alimentaires en cas d’impayés.

Enfin, nous sommes plusieurs dans cet hémicycle à défendre un principe qui nous tient particulièrement à cœur, madame la ministre, celui de la solidarité fiscale, une violence économique peu visible, mais bien réelle. Il n’est pas concevable qu’une femme, bien que divorcée, continue à être solidairement responsable des dettes contractées par son conjoint, sans son consentement. Ces femmes aussi ont besoin de nous avoir à leurs côtés, et notre société s’honorerait à leur apporter des réponses concrètes ! La parole

Nous démarrons l’examen de ces crédits dans un contexte très particulier, vous le savez, un contexte difficile pour notre pays,

C’est un enjeu d’avenir, un enjeu de souveraineté qui doit guider l’ensemble de la représentation nationale et, évidemment, du Gouvernement. Dans ce contexte particulièrement difficile sur le plan économique, les crédits alloués à la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » sont non seulement préservés, mais connaissent

pour préserver nos politiques de solidarité. Je salue à cet égard la position des groupes qui ont annoncé apporter leur soutien à l’adoption des crédits Sans être exhaustive, permettez moi de mentionner plusieurs composantes majeures de ce budget : le respect des engagements du pacte des solidarités avec la tarification des cantines à 1 euro et le programme Mieux manger pour tous, les crédits dédiés à la lutte contre la précarité

le préremplissage des demandes de prime d’activité et de RSA, afin que chacun dispose du niveau de soutien adéquat, que ce soit à la hausse ou à la baisse, lorsque des indus sont détectés.

le programme 157 « Handicap et dépendance », en hausse de 650 millions d’euros, je tiens à souligner la montée en charge de la déconjugalisation de l’AAH, qui représente un gain moyen pour les nouveaux bénéficiaires de 556 euros par mois, supérieur aux 370 euros initialement estimés.

pour explication de vote.

avec un temps partiel, au delà de 50 %. Il est très important de maintenir ce dispositif, qui affecte très directement la vie quotidienne des personnes en situation de handicap qui travaillent.

de poursuivre une activité tout en continuant à percevoir l’allocation. L’année dernière, cette mesure n’a été que partiellement mise en œuvre, faute d’avoir été préparée par les administrations.

Ce rapport a été publié en février 2024. Il conclut que la reconduction du Fatésat suppose « une meilleure évaluation de l’utilisation des crédits et de leur impact sur l’activité économique des Ésat que la consolidation de la résilience économique des Ésat constitue un préalable à tout dispositif d’aide spécifiquement axé sur le secteur. Toutefois, il n’est pas impossible que la reconduction du Fatésat permette précisément de consolider la résilience économique des Ésat.

dans le cadre du programme de contrôle de la commission des finances pour l’année 2025, Pierre Barros et moi même avons souhaité nous consacrer à l’évolution du financement des violences faites aux femmes, au premier rang desquelles figure évidemment le système prostitutionnel.

dispositions proposées par notre collègue Laurence Rossignol et les autres membres du groupe socialiste, ainsi que les amendements précédents, d’ailleurs, posent en creux la question des moyens nécessaires pour lutter contre les violences faites aux femmes. Je l’ai dit dans mon intervention générale, les moyens de l’État en faveur de l’égalité femmes hommes, singulièrement lutte contre les violences faites aux femmes, sont largement insuffisants. L’affaire Gisèle Pelicot a révélé l’omerta qui persiste sur les violences intraconjugales. de cette macabre histoire, de nombreux témoignages de victimes ont surgi grâce au courage de cette femme. Le Gouvernement doit être à la hauteur des attentes de la société pour lutter contre les violences

sociale et physique ayant pour effet de diminuer la capacité d’action de la victime et de provoquer un état de vulnérabilité doivent effectivement être reconnues comme des violences psychologiques.

constitue une avancée essentielle. Cependant, l’efficacité de ce dispositif dépend largement du soutien et de l’accompagnement fournis par le réseau associatif. En effet, ce sont les associations, par leur expertise et leur engagement, qui permettent de maximiser l’impact du TGD, en assurant un suivi des bénéficiaires et en les aidant à retrouver leur autonomie. Dans cette perspective, il semble impératif d’augmenter les subventions attribuées aux associations. Selon les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), l’accompagnement d’une personne détentrice d’un TGD représente un coût moyen de 1 200 euros par an. Ce montant couvre les services de soutien émotionnel, juridique et social qui sont nécessaires pour que la victime puisse se sentir en sécurité. À l’heure actuelle, environ 6 000 TGD sont déployés en France, ce qui entraîne un besoin important de ressources pour les associations qui accompagnent

Toutefois, je ne me souviens pas avoir été alerté sur la nécessité de déployer en urgence 1 500 TGD supplémentaires. Si ce besoin existe, nous sommes prêts à y répondre.

ce qui représente un taux de réponse de 86 %, en nette progression par rapport aux années précédentes – cela signifie aussi que presque 15 % des appels n’ont pas reçu de réponse. Pour 2025, l’objectif est d’atteindre un taux d’appels traités de 95 %. mes chers collègues, il est difficile d’imaginer que 5 % des appels de femmes victimes de violence demeurent sans réponse. C’est pour cette raison que nous vous proposons d’augmenter les moyens de cette plateforme. Quel

Mikaele Kulimoetoke. Il s’agit d’un amendement d’une importance capitale pour ma petite collectivité de Wallis et Futuna.

qu’avec des bénévoles et elle estime ses besoins à 415 000 euros. Cette structure pourra améliorer la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences, notamment en facilitant l’accès à un hébergement d’urgence dans un bâtiment mis à disposition qui a encore besoin de travaux. Cette dotation servira de surcroît à fournir un accès à des soins psychologiques et à assurer la formation des intervenants locaux, afin de sensibiliser les jeunes générations. Cette association existe depuis une dizaine d’années et fonctionne avec des moyens notoirement insuffisants. Nous le savons tous, mes chers collègues, il est difficile de demander de l’aide, d’autant plus lorsque le territoire compte

Dès lors, la Fédération des acteurs de la solidarité, aux côtés de ses partenaires spécialisés, demande que, dans le cadre du nouveau plan interministériel pour l’égalité entre les femmes

je rappelle que je conduirai cette année, avec notre collègue Pierre Barros, un contrôle budgétaire sur l’évolution du financement de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les conclusions de ces travaux seront évidemment publiques, si la commission des finances le veut bien. En attendant, je réitère ma demande de retrait de cet amendement.

Plus encore, il faut agir financièrement pour accompagner associations et départements. C’est la raison pour laquelle nous avons proposé de financer ce plan d’urgence pour les pouponnières. Quel est l’avis de la commission ?

et la sécurité sociale. Si la stagnation de leurs capacités d’accueil est en effet de plus en plus inquiétante, l’ajout d’un nouveau financement de l’État, qui plus est à un montant aussi élevé, risquerait d’ajouter à la complexité de la gouvernance du secteur médico social. J’ajoute que le PLF pour 2025 contient déjà plusieurs mesures de soutien direct aux départements, notamment la possibilité d’augmenter le taux des droits de mutation à titre onéreux Ces mesures me semblent préférables aux dotations de l’État, puisqu’elles valorisent l’autonomie et la responsabilité des collectivités au travers de leurs ressources propres et le libre exercice de leurs compétences. La commission émet donc un avis défavorable. Quel est l’avis du Gouvernement ?

dans la lutte contre la pédocriminalité ; garantir des soins spécifiques. Aujourd’hui, il est impératif de mettre en place une stratégie nationale pour prendre en charge les psychotraumatismes causés aux enfants par les violences sexuelles et intrafamiliales. Cet amendement vise à répondre à cette nécessité. Quel est l’avis de la commission ?

Ces questions devraient donc être laissées aux départements, au plus proche du terrain, et à la sécurité sociale dans le cadre du débat sur les PLFSS. Je ne reviens pas sur ce que j’ai dit précédemment

enfance. La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi Taquet, constitue une avancée, puisqu’elle dispose que « les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité », sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur

Par ailleurs, nous avions obtenu ici même, l’année dernière, que le Gouvernement augmente de 32 millions d’euros les financements de la prise en charge des mineurs non accompagnés.

enfants en danger (Uaped) sont encore trop peu connues du grand public, alors qu’elles jouent un rôle immense en matière de protection de l’enfance. Les équipes de ces unités d’accueil

soit une par juridiction. Mes chers collègues, derrière chaque chiffre, il y a des vies d’enfants que nous devons protéger, des enfants dont l’espérance de vie est amputée de vingt ans en moyenne lorsqu’ils subissent des violences intrafamiliales violences est évalué à 38 milliards d’euros par an, soit 1,4 % du PIB. Pourtant, alors que 21 nouvelles unités étaient prévues en 2024, seules 17 ont pu être financées pour 2025. Bien que 4 millions d’euros soient inscrits dans le PLFSS pour l’ouverture de 25 nouvelles unités, les crédits destinés à la coordination des professionnels intervenant dans ces structures, qui figurent dans le programme 304 de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances d’euros. Par cet amendement, mon collègue Xavier Iacovelli propose donc d’abonder de 4 millions d’euros supplémentaires les crédits du programme 304, afin d’aligner les moyens de coordination des équipes de soignants sur le rythme d’ouverture de ces unités. Cette

je le rappelle,

quel que soit leur secteur d’activité. Cet accord a été signé entre les partenaires sociaux de la branche, salariés et employeurs, et a été homologué par le Gouvernement peu de temps après. Néanmoins, nombreux sont les gestionnaires inquiets de la situation résultant de cet accord. Nos auditions nous ont montré que certains organismes sont réticents ; ils refusent même d’affecter la bonne enveloppe au financement desdites revalorisations, car le versement des primes Ségur met en péril leur équilibre financier. Sur ce point, l’avis de la commission est nuancé. Sur le principe, nous relevons que la situation dans laquelle nous nous trouvons n’est guère orthodoxe, puisqu’il reviendrait à l’État de financer la politique salariale d’une branche particulière. La commission a notamment relevé que ces deux amendements, ainsi que ceux qui suivent, ne visent pas les mêmes structures

d’appliquer cette mesure, et ce sans compensation. Les membres de cette assemblée savent bien dans quel état sont les finances des collectivités.